La séance est reprise. Monsieur le ministre, mes chers collègues, M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre communication du décret de M. le Président de la République en date du 27 juin 2018

Par lettre en date de ce jour, le Gouvernement a demandé l'inscription à l'ordre du jour du lundi 2 juillet, après-midi et soir, de la suite de l'examen du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Acte est donné de ces modifications.

est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au et figurera dans l'analyse politique du scrutin. Nous reprenons l'examen du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

est à Mme la rapporteur. Cet amendement tend à revenir sur la concurrence déloyale de certaines productions étrangères qui, bien que commercialisées en France, ne respectent pas les normes européennes et françaises imposées par ailleurs à nos agriculteurs, du point de vue tant des traitements que des modes de production. Sont en particulier visés le traitement par des produits phytopharmaceutiques dont l'usage est interdit en France et dans l'Union européenne, l'utilisation des antibiotiques comme activateurs de croissance, l'inclusion de farines animales dans l'alimentation des bovins ou encore le non-respect des normes environnementales ou des exigences d'identification et de traçabilité. Au-delà de la distorsion de concurrence qu'elles engendrent pour nos agriculteurs, ces importations de denrées ou de produits constituent une menace tant pour la santé publique que pour l'environnement. Il importe donc d'assurer l'effectivité d'interdictions certes déjà posées par le droit européen et français, mais que certains produits importés parviennent aujourd'hui à contourner. Le présent amendement vise en outre, monsieur le ministre, les moyens dédiés au contrôle de ces normes par les services des douanes et de la répression des fraudes, afin qu'ils puissent mener des campagnes de contrôle plus massives, plus régulières et donc plus fiables d'exiger systématiquement, dans chaque accord de libre-échange, la possibilité de faire des contrôles, car bon nombre de pratiques ou de traitements ne sont plus décelables à la réception des produits en France ; enfin, de mettre en oeuvre systématiquement des clauses de sauvegarde pour suspendre l'importation de telle ou telle production

Mme Nicole Bonnefoy. Cet amendement, que nous avons déjà proposé en commission, vise à interdire l'importation, la vente ou la distribution à titre gratuit de denrées alimentaires traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant des résidus de substances actives non autorisées par les autorités communautaires. Il s'agit de préserver la santé de nos concitoyens, tout en luttant aussi contre les distorsions de concurrence entre producteurs européens et non européens.

pour interdire la commercialisation en France de cerises traitées avec ce produit. Cet amendement tend donc à généraliser ce principe, sans avoir à passer par une décision gouvernementale, parce qu'il n'est plus acceptable que nous puissions avoir sur notre marché des denrées traitées avec des produits que nous savons dangereux pour la santé humaine

entre les producteurs européens et les producteurs des pays tiers, tout en protégeant la santé publique et l'environnement. Certaines molécules chimiques interdites en Union européenne sont pourtant utilisées

l'Atrazine, interdite dans l'Union européenne depuis le début des années 2000. Une telle situation n'est pas tenable pour les agriculteurs français dont les produits agricoles doivent respecter des pratiques agricoles plus coûteuses et qui se trouvent concurrencés par ceux de producteurs étrangers ayant des contraintes environnementales moindres.

Lors des contrôles effectués en 2014, un total de 3 265 échantillons a dépassé ces limites, dont la grande majorité était des produits importés. Parmi ceux-ci, 1 253 contenaient des pesticides non autorisés par l'Union européenne. Or, ces dernières années, selon les statistiques des douanes, seulement une poignée de produits ont été interdits. C'est pourquoi, tout en continuant d'aller dans la voie de la réduction des produits phytosanitaires, il est nécessaire d'arrêter l'importation de produits qui ont été traités par des molécules interdites en France.

Il s'agit de ne pas introduire de distorsion de concurrence, je l'ai dit- nos producteurs y sont extrêmement sensibles, et cela se comprend tout en protégeant la santé publique et l'environnement. Nous avons déjà évoqué cette question à de nombreuses reprises. Nous pouvons faire tous les efforts possibles pour tenter de répartir la valeur et de mieux rémunérer nos producteurs, mais, tant que nous serons soumis à un commerce international dérégulé, nos efforts seront en partie sans effet. Notre agriculture, à laquelle nous tenons tous, est exposée à la concurrence de denrées produites dans des conditions qui n'ont rien à voir avec celles qui se pratiquent dans notre pays, au point de tant social que sanitaire et environnemental. Ce n'est acceptable ni pour les consommateurs ni pour les producteurs. Il s'agit aussi de ne pas favoriser ces modes de production dans les autres pays du monde. Chaque région, plutôt que de s'engager dans une course au moins-disant et de développer des filières d'exportation à grand renfort d'intrants et de phytosanitaires, doit retrouver une souveraineté alimentaire ; qu'on se l'applique aussi

produits phytopharmaceutiques, farines animales ou encore antibiotiques activateurs de croissance. Il s'agit de ne pas laisser subsister de distorsion de concurrence entre les producteurs européens et les producteurs des pays tiers, tout en protégeant la santé publique et l'environnement. Le rapport de la commission Schubert sur les impacts du CETA répertorie les activateurs de croissance et les produits phytosanitaires- -interdits dans l'Union européenne mais autorisés dans les produits exportés vers l'Union européenne, comme l'Atrazine, interdite dans l'Union depuis le début des années 2000. Une telle situation n'est pas tenable pour les agriculteurs français, dont les produits agricoles doivent respecter des pratiques plus coûteuses et qui se trouvent concurrencés par ceux de producteurs étrangers ayant des contraintes environnementales moindres. Tel est l'objet de cet amendement.

qui ne respectent pas les normes européennes et françaises, en matière de traitement, pour les premiers amendements, ou de mode de production, pour les deux derniers. Nous l'avons dit, ces préoccupations sont légitimes, mais elles sont intégralement satisfaites

est quelque chose que l'on porte à l'échelon européen, et cela fait partie de la feuille de route sur la sortie et la réduction des pesticides que le Gouvernement soutient. Nous travaillons sur la sortie des produits au fur et à mesure que nous avançons dans nos travaux.

les dispositifs d'évaluation européenne, accélérer la sortie des molécules les plus préoccupantes vis-à-vis de l'Union européenne, je viens de le dire, diminuer la quantité de pesticides utilisés, revoir la redevance pour pollution diffuse en ciblant les substances les plus préoccupantes, mais aussi mieux connaître les impacts pour informer et protéger notre population et l'environnement. Donc, là aussi, nous misons sur la recherche

recours aux préparations naturelles peu préoccupantes, tout en préservant, évidemment, une évaluation sanitaire et environnementale préalable. Cela passe par le développement de la formation, par la réorganisation du conseil, par les stratégies et les plans de filière ; n'oublions pas que, dans tous les plans de filière qui nous ont été adressés- plus de trente-cinq -, il y a des engagements,

qu'à ce niveau. Je souhaite rappeler que les denrées alimentaires d'origine animale importées sont soumises à un contrôle sanitaire lors de leur introduction sur le territoire de l'Union européenne, et peuvent ensuite circuler librement entre les États membres dans le cadre du marché unique. Prendre une telle mesure en droit français, d'une part, ne serait pas efficace parce que, vous le savez comme moi, il y a des produits qui entrent par d'autres États membres, sur lesquels on appose un beau logo «

les concessions commerciales de l'Union européenne à des garanties relatives au mode de production, y compris en matière de promoteurs de croissance et de traçabilité, et à les inscrire dans les limites soutenables pour les filières en cause. C'est ce que nous faisons sur les accords commerciaux.

ne soient pas issues d'animaux ayant reçu des antibiotiques comme promoteurs de croissance. C'est un enjeu de santé publique, car les antibiotiques délivrés comme tels concourent au développement de l'antibiorésistance. Cet accord a été obtenu par le Parlement et par le Conseil

Donc, un peu de cohérence, un peu de motivation, et allez-y, nous serons derrière vous

s'ils se présentent dans un élevage et qu'un animal n'a aucune boucle, celui-ci va à l'équarrissage. Or il y a aujourd'hui des importations de viande

c'est un grand pas, mais nous nous réjouirons encore davantage de la mise en application rapide de cette décision. Il ne faudrait pas que la Commission mette trois ans à publier les règlements d'application. Je suis d'accord. Donc nous comptons sur vous pour que ce dispositif s'applique rapidement et puisse s'imposer dans le cadre des traités de libre-échange CETA, MERCOSUR et tous les autres.

et c'est votre responsabilité, monsieur le ministre, de taper du poing sur la table, de ne pas vous laisser tondre la laine sur le dos, comme on dit en pastoralisme. Cela relève aussi de l'Europe. Vous avez un double travail,

Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier mes collègues de la commission des affaires économiques qui ont eu la clairvoyance d'insérer un alinéa 6 à l'article 11 . Ainsi, Ainsi, serait intégré aux missions de la politique agricole et alimentaire le fait de « s'assurer dans tout nouvel accord de libre-échange d'une réciprocité effective [ ...], d'une exigence de normes de production comparables, ainsi que d'un degré élevé d'exigence dans l'élaboration de normes communes sanitaires et phytosanitaires [ ...] en vue d'une protection toujours plus forte des consommateurs et d'une préservation de nos modèles agricoles européens ». Cela est particulièrement vital pour nos agriculteurs, nos concitoyens et nos modèles agricoles, au regard de la frénésie de l'Union européenne à négocier et à conclure des accords de libre-échange nouvelle génération avec des pays tiers- MERCOSUR, Indonésie, Mexique, Chili -, sachant par ailleurs que les négociations avec Singapour en 2014, le Vietnam en 2016 et le Japon en décembre 2017 sont closes. Or ces nouveaux accords affectent de manière profonde l'économie des pays signataires, dans la mesure où ils ne se contentent pas de lever les barrières tarifaires. On reproche d'ailleurs à la Commission européenne de mener une politique commerciale déséquilibrée, qui prend insuffisamment en compte une exigence de réciprocité de la part des partenaires. Cette question concerne particulièrement l'ouverture des marchés publics, mais aussi les procédures et les normes sanitaires et phytosanitaires, au détriment des agriculteurs européens, dont les agriculteurs français que nous défendons ici. Je prends pour exemple l'accord UE-MERCOSUR, qui aurait des conséquences importantes sur nos populations, de manière directe et indirecte. Tout d'abord, il constitue un véritable désastre pour la sauvegarde de l'environnement pour la sauvegarde de l'environnement et du climat- l'élevage bovin brésilien est responsable, à lui seul, de 80 % de la destruction de la forêt amazonienne. les exportations de viandes et de volailles prévues dans l'accord sont particulièrement inquiétantes, car les mesures sanitaires et phytosanitaires dans ces pays ignorent le principe de précaution et permettent de nourrir avec des OGM les animaux et les volailles, en plus de les soumettre aux piqûres aux hormones de l'Union européenne, de 100 000 tonnes de boeuf et de 90 000 tonnes de volaille, ainsi qu'un quota total de 600 000 tonnes de canne à sucre. On voit donc bien tout l'intérêt de cet article.

sur un aspect spécifique de cet article, à savoir l'alinéa qui prévoit que la politique agricole favorise, pendant l'enfance et l'adolescence, l'acquisition d'une culture générale de l'alimentation. Je souhaite prendre la parole sur ce thème, car deux de mes amendements sur ce sujet ont été déclarés irrecevables. Le premier prévoyait la mise en place obligatoire, dans les écoles, d'un jardin pédagogique. Le second, pour échapper à l'article 40 de la Constitution, visait à favoriser cette pratique dans le cadre de l'éducation à l'alimentation. Je pense que ces mesures auraient eu toute leur place dans ce texte. Si l'on veut favoriser une alimentation durable, des comportements alimentaires sains, des jardins pédagogiques ont toute leur importance. C'est un outil utile pour la sensibilisation et l'éducation à l'alimentation. Il permet aux élèves de redonner une valeur à leur alimentation, d'être sensibilisés au gaspillage alimentaire, au traitement des déchets la mise en place de compost. Il permet une forme de reconnexion à la nature. Aujourd'hui, ces enseignements sur l'agronomie, la botanique, les sciences de la vie et de la terre, ou SVT, sont de plus en plus rares. Les SVT ont été l'une des grandes perdantes de la réforme du baccalauréat. Nous perdons ainsi une culture essentielle à notre bien-être ! Les agriculteurs se plaignent de ne pas être compris par le reste de la population. Il serait crucial d'avoir une éducation dès le plus jeune âge dans ces domaines.

Pour favoriser les importations de ces produits, l'Union européenne a relevé ses seuils, à l'inverse de ce qui se fait en France. Ainsi, depuis 2012, les lentilles canadiennes ou américaines peuvent entrer sur le territoire européen pour être consommées avec un taux

différente, vise à interdire l'importation en France de denrées produites en utilisant des substances interdites dans l'Union européenne et en France, même à doses résiduelles : produits phytopharmaceutiques, farines animales, antibiotiques, activateurs de croissance

Face à cette incohérence, il est légitime que les agriculteurs ressentent une profonde injustice. Avec le CETA, des milliers de tonnes de volaille, de viande porcine ou bovine ou de sucre vont inonder le marché communautaire. La France, signataire de cet accord, va ainsi importer des marchandises produites avec des molécules qu'elle interdit. En effet, le rapport de la commission Schubert sur les effets du CETA répertorie des activateurs de croissance et des produits phytosanitaires-

Une telle situation n'est pas tenable pour les agriculteurs français, dont les produits agricoles doivent respecter des pratiques plus coûteuses et qui se retrouvent concurrencés par ceux de producteurs étrangers dont les contraintes environnementales sont moindres. La parole

L'objectif est d'empêcher des distorsions de concurrence entre les producteurs européens et ceux des pays tiers, tout en protégeant l'environnement et la santé publique. Une telle situation n'est pas tenable pour les agriculteurs français, dont les produits agricoles doivent respecter des pratiques plus restrictives,

dans la politique de l'alimentation. Cela permettra d'assurer une cohérence avec les modifications apportées par le projet de loi au programme national nutrition santé et aux programmes alimentaires nous proposons de remplacer l'aide alimentaire par la lutte contre la précarité alimentaire dans les objectifs de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation.

aux farines animales dans des, sont parfaitement incompatibles avec le modèle d'élevage prôné par les États généraux de l'alimentation et les objectifs de la politique de l'agriculture et de l'alimentation définie au livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime. Cette pratique, strictement interdite au sein de l'Union européenne, ne fait aujourd'hui l'objet d'aucune restriction pour les importations affirmer que toute viande entrant sur le marché européen respecte les mêmes normes de production que celles qui sont imposées aux producteurs communautaires est donc mensonger. Elle soulève, en outre, des questions de santé publique : alors que l'utilisation des farines animales dans l'alimentation des bovins a été strictement prohibée en Europe, à la suite de la crise de la vache folle, il semble à la fois incohérent et risqué d'autoriser des importations de viandes issues de bovins ayant consommé de telles substances. C'est pourquoi cet amendement vise à renforcer le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, en exprimant clairement le refus de la France d'importer des viandes bovines issues d'animaux nourris aux farines animales.

n° 244 rectifié . Nous proposons que la France refuse d'importer des viandes issues de bovins engraissés aux antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance.

le Gouvernement s'est engagé à défendre le modèle européen de production agricole dans les enceintes internationales et dans l'ensemble des négociations commerciales de l'Union européenne. Ainsi, nous conditionnons les concessions commerciales de l'Union européenne

Il s'agissait pour nous de faire préciser dans la loi que tout accord de libre-échange doit s'appuyer sur l'exigence de normes de production comparables entre les pays de l'Union européenne et les pays tiers. L'objectif est d'assurer la qualité des produits destinés aux consommateurs européens, tout en protégeant nos agriculteurs d'une concurrence qui pourrait s'avérer déloyale.

à étendre le champ des normes pour lesquelles l'exigence de réciprocité doit s'appliquer, en intégrant celles qui sont relatives au bien-être animal. Nous voterons donc l'amendement rédactionnel du Gouvernement, qui appuie la position prise depuis plusieurs années par le Sénat sur la question des accords de libre-échange. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

Celle-ci est essentielle, notamment pour la fertilité, la régulation du cycle de l'eau, la lutte contre l'érosion, ou encore la santé des plantes. Le sol représente 80 % de la biomasse. Cette biodiversité complexe et essentielle a une valeur, a une valeur, tant pour la qualité de notre environnement, que pour la production agricole. L'érosion des sols est un phénomène qui s'accentue et qui est inquiétant, à la fois pour la baisse des rendements agricoles, mais aussi pour les phénomènes de ruissellement et d'inondation qui peuvent être provoqués par un sol quasi mort,

Il convient donc de préciser que la protection et la valorisation des terres agricoles impliquent une protection de la biodiversité des sols. J'en profite pour présenter un amendement jugé irrecevable. Il portait sur la protection de la quantité quantité des sols, non moins importante que leur qualité. Cet amendement avait pour objet de donner une valeur législative à l'engagement du Gouvernement en matière de lutte contre l'artificialisation des sols. C'était un cavalier ! Nous perdons 236 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers par jour, ce qui correspond à la consommation d'un département français tous les sept ans. Cette artificialisation se fait majoritairement

je vous remercie

un sol fertilisé, riche en matières organiques, donc en carbone, permet de mieux résister à l'érosion et de lutter contre les inondations.

La France et l'Union européenne souffrent d'une dépendance en protéines végétales historique, issue en grande partie des accords commerciaux négociés dans le cadre du GATT dans les années 1960. On ne le répète jamais assez. La France est dépendante en ce domaine à plus de 40 européen global est encore plus fort. Or cette dépendance en protéines végétales pose de nombreux problèmes. Elle soumet notamment les éleveurs français qui dépendent d'importations pour l'alimentation animale à la volatilité des cours mondiaux dans un contexte international tendu.

présentent des avantages sur les plans agronomique et environnemental. Par exemple, le développement des légumineuses permet l'enrichissement des sols en azote. Introduire du soja dans les rotations permet aussi de limiter les intrants. Des filières commencent à se développer et la politique agricole doit les encourager. L'autonomie protéique est souhaitable à la fois sur le plan de la sécurité alimentaire et d'un point de vue économique, social et environnemental. Cet objectif est stratégique

Quel plan Protéines pour l'Europe ? Plus ça ira, plus nous serons dépendants en matière de protéines végétales. Je pense plus particulièrement aux légumineuses. Pour avoir été moi-même président de l'interprofession française et européenne des protéines, je sais les difficultés pour développer cette filière. S'il n'y a pas une volonté politique d'accompagner le développement de la recherche génétique sur des plantes riches en protéines, nous n'aboutirons pas et nous serons de plus en plus vulnérables et dépendants du reste du monde.

Quelle ambition avons-nous ? Il y a un vrai problème. Vous dites vouloir marquer l'histoire de la France par une reconquête, un renouveau de l'agriculture, avec une nouvelle stratégie permettant une meilleure indépendance et une meilleure traçabilité de l'alimentation répondant aux attentes des citoyens.

Les potagers et jardins pédagogiques permettent une appropriation douce de la nature et favorisent la prise de conscience de la biodiversité dès le plus jeune âge. Les élèves qui ont la chance de cultiver des fruits et des légumes tout au long de l'année seront sensibilisés à la fois au respect de l'environnement et à une alimentation saine. Pour rappel, en novembre 2016, un appel à projets « Potagers et jardins pédagogiques » avait été lancé par le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer. Il y avait eu alors plus de 10 000 manifestations d'intérêt, et plus de 1 300 établissements avaient été désignés lauréats de cette opération. Plusieurs d'entre eux font aujourd'hui la promotion de cette expérience, riche d'enseignements pour les élèves. L'éducation à l'alimentation et au développement durable est un levier majeur pour faire évoluer les comportements. C'est dès le plus jeune âge qu'il faut éclairer le consommateur en devenir pour relever les défis de la transition écologique et de la santé publique. C'est aussi une expérience qui a du sens et qui donne un nouveau souffle au projet global d'alimentation saine et durable. J'irai plus loin pour clore mon propos : ce seront des graines favorables semées dans la tête de nos enfants, initiés non seulement au goût d'aliments qu'ils auront eux-mêmes cultivés, mais aussi à de futures pratiques responsables.

Et son corollaire : quels enfants allons-nous laisser à notre planète ? L'éducation à l'environnement, l'éducation à l'alimentation, l'éducation à la citoyenneté : tout est lié

Guillaume Gontard. Cet amendement a pour ambition de donner les moyens à la politique nationale de l'alimentation d'atteindre les objectifs de transition qu'elle s'est fixés en matière de restauration collective. Un de ces moyens est la création d'un « bonus cantines bio et locales Le passage à 20 % ou même à 30 % de bio n'entraîne pas nécessairement de surcoûts pour les établissements publics, mais une politique plus ambitieuse peut, en fonction des territoires et dans un premier temps, nécessiter un budget supplémentaire, notamment pour des besoins de formation ou de matériel. Nous souhaitons donc créer un « bonus cantines bio et locales » pour accompagner clairement la transformation de la restauration collective à travers un montage de financements publics et privés. Ce dispositif doit continuer à être travaillé dans le cadre des réflexions sur le financement de la transition agricole et alimentaire, notamment le volet alimentation des dispositifs de financement prévus par les Nous avons eu un débat hier sur l'intérêt pédagogique de favoriser le bio et le lien avec la provenance des aliments. La question des jardins pédagogiques abordée par Joël Labbé et Angèle Préville est aussi très intéressante. Pour mener à bien ces projets, les collectivités doivent être accompagnées et aidées. C'est le sens de cet amendement. Les

encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. À cette fin, il préconise des actions pour favoriser l'approvisionnement de la restauration collective, publique comme privée, en produits agricoles de saison ou en produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine, notamment issus de l'agriculture biologique. Par le biais de cet amendement, nous souhaitons aller plus loin en soutenant les collectivités et les établissements les plus fragiles situés en zone urbaine ou rurale dans la transition agricole et alimentaire. Il est de notre devoir de faciliter la mise en oeuvre volontariste des mesures d'adaptation de la restauration collective à une alimentation qualitative. C'est la raison pour laquelle il paraît indispensable d'accompagner financièrement les collectivités qui en ont particulièrement besoin. Tel est l'objet de cet amendement.

l'Union européenne et l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay, est en effet source d'inquiétudes pour les agriculteurs et les consommateurs. Les différences de réglementation entre nos deux continents semblent menacer notre système agricole d'une concurrence peu loyale. Le cas des importations de viande bovine est régulièrement évoqué. Cet accord entraînerait l'importation de 70 000 tonnes de viande bovine sud-américaine chaque année. Ces nouvelles importations auront un effet direct et immédiat sur la filière bovine française et européenne. Il est donc important de conduire ces négociations internationales en ayant à l'esprit leurs incidences concrètes. En outre, cette substitution de certains produits agricoles étrangers aux produits agricoles européens doit se faire sous des conditions de respect de nos critères sanitaires. Il faut donc établir des procédures de traçabilité du produit et de certification sanitaire, afin d'évaluer la qualité nutritionnelle et hygiénique de l'alimentation des consommateurs européens. Le scandale, en mars 2018, du poulet brésilien avarié, mais aussi la présence de salmonelle dans les exportations du géant BRF mis en évidence les risques des accords d'importation de viande sud-américaine. La police brésilienne avait en effet mis au jour un réseau d'inspecteurs d'hygiène corrompus qui certifiaient de la viande avariée comme propre à la consommation. La parole est à M. Bernard Delcros, pour défendre

entre l'Union européenne et le Canada, le CETA, sur l'environnement, le climat et la santé. Cette commission a rendu ses conclusions à l'automne dernier, conformément à ce qui avait été demandé. Cela a donné lieu à un plan d'action du Gouvernement sur la mise en oeuvre du CETA. du CETA. En cours de négociation, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les quatre pays du MERCOSUR inquiète à son tour agriculteurs et associations de consommateurs. En cause, les différences de réglementation entre les deux régions qui font peser la menace d'une concurrence peu loyale entre les producteurs européens et ceux Par exemple, les farines animales ou l'utilisation d'antibiotiques comme activateurs de croissance sont autorisées dans les pays du MERCOSUR, mais interdites dans l'Union européenne. De même, alors que cet accord pourrait conduire à l'importation de près de 70 000 tonnes de viande bovine sud-américaine par an, il est fondamental de s'interroger en amont sur les procédures de traçabilité et de certification sanitaire pratiquées dans cette région, afin que cet accord n'ait pas des effets préjudiciables à la qualité nutritionnelle et sanitaire de l'alimentation des consommateurs européens. Aussi, nous demandons au Gouvernement de nommer, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, une commission d'experts indépendants sur le modèle de la commission Schubert. lui remettra, dans un délai d'un an, un rapport sur les effets économiques, sociétaux et sanitaires qu'aurait la ratification de l'accord de libre-échange avec les pays du MERCOSUR pour la filière agricole, ainsi que sur les risques liés à la dégradation de la qualité alimentaire, notamment en raison des différences de normes d'hygiène potentiellement existantes.

Les MAE consistent en des contrats sur cinq ans, qui tendent à définir et encourager des pratiques agricoles spécifiques, respectueuses de l'environnement. Les agriculteurs qui les mettent en oeuvre peuvent alors percevoir un montant majoré d'aides Ces crédits sont cadrés par le règlement européen, dit agroenvironnemental, du 30 juin 1992. Chaque État membre en a subsidiairement fait sa propre déclinaison. La manière dont la France décline aujourd'hui sa stratégie agricole est fondée sur une logique de moyens, et non d'objectifs.

Le rapport demandé dans cet amendement permettrait de préciser les objectifs poursuivis avec les MAE, dans le cadre de la stratégie globale de la France en matière agroenvironnementale, et d'analyser dans quelle mesure les moyens mis en oeuvre conduisent aux buts visés.

pour la mise en oeuvre des MAE au titre du FEADER, doivent déjà établir des rapports annuels de mise en oeuvre, aussi appelés RAMO, où sont renseignés les différents indicateurs de réalisation. Pour ces raisons, je suis défavorable à cet amendement.

Cet article consacre la mention « haute valeur environnementale », ou HVE, en lui conférant une définition législative et en la liant aux démarches agroécologiques. Il s'agit de privilégier les modes de production agroécologiques, c'est-à-dire une façon de concevoir des systèmes de production qui s'appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. L'agroécologie implique le recours à un ensemble de techniques qui considèrent l'exploitation agricole dans son ensemble. C'est grâce à cette approche systémique que les résultats techniques et économiques peuvent être maintenus ou améliorés tout en renforçant les performances environnementales. L'agroécologie réintroduit de la diversité dans les systèmes de production agricole et restaure une mosaïque paysagère diversifiée ; le rôle de la biodiversité comme facteur de production en sort renforcé, voire restauré.

Cet article précise la définition législative de la mention « haute valeur environnementale » en la liant à la démarche agroécologique. Près de dix ans après sa création, cette notion valorisante n'a malheureusement presque pas été utilisée. Comme nous l'avons expliqué lors de la défense d'un précédent amendement, elle présente pourtant un réel intérêt, notamment lorsqu'on atteint le niveau 3 de certification, qui s'accompagne du respect d'indicateurs de performance. Cet amendement tend donc à donner un nouveau souffle à la en en faisant une mention valorisante de l'agroécologie. Aujourd'hui, alors même que celle-ci est admise par tout le monde, elle ne bénéficie pas d'un label qui lui soit spécifique. Il s'agit par conséquent de prévoir un label public qui permettrait de certifier la démarche agroécologique des exploitants agricoles. Bien évidemment, il n'est pas question d'en faire le seul label. Nous sommes d'une manière générale favorables au soutien de toutes les certifications, qui, à l'instar des labels ou mentions valorisantes, participent à la montée en gamme de notre agriculture.

c'est limiter les engrais de synthèse, c'est réduire les produits phytosanitaires, c'est préserver l'eau et l'énergie, et ce sont des performances économiques, sociales et environnementales.

que beaucoup de américains s'étaient engagés dans des démarches de certification quasiment de type ISO. Je suis convaincu que, en tant

il est absolument évident que les agriculteurs, quels qu'ils soient, contribuent à l'entretien de l'environnement, parce que c'est la base fondamentale de leur métier. Cela étant dit, certains d'entre eux se sont lancés dans des démarches expérimentales

? Les États généraux de l'alimentation ont réaffirmé la nécessité de prendre davantage en compte les questions relatives à l'environnement et de concilier la performance économique et la performance environnementale.

vise à encadrer la définition de la certification « haute valeur environnementale » pour les produits issus de l'élevage et à imposer de nouvelles obligations en matière d'exigence de résultats. La certification HVE est aujourd'hui très majoritairement utilisée par des exploitations végétales ou vitivinicoles. Or il est essentiel que les éleveurs puissent prétendre à une certification qui prenne en compte des enjeux environnementaux environnementaux et nutritionnels. C'est la raison pour laquelle nous proposons que soient fixés par décret de nouveaux critères de définition de la pour l'élevage sur une base d'obligation de résultat. Les objectifs seraient la diminution des émissions de gaz à effet de serre, l'amélioration de la qualité nutritionnelle des produits animaux et la diminution de la déforestation importée. J'ai noté, monsieur le ministre, votre soutien

La question de l'adaptation de la certification environnementale aux élevages d'animaux a été soulevée au cours de nos auditions. Il est néanmoins apparu qu'il existait déjà quelques élevages certifiés. Cette notion mérite certainement des éclaircissements de la part du Gouvernement, notamment au regard des travaux qui seraient en cours sur ce sujet.

Madame la sénatrice, la HVE est une certification d'exploitation et non pas une certification de filière. On ne peut donc pas définir des exploitations Les indicateurs de performance qui identifient les exploitations bénéficiant de ce label seront revus dans le cadre des travaux de la Commission nationale de la certification environnementale, afin de mieux

Cette garantie est importante pour le consommateur, ainsi que pour les professionnels qui interviennent dans l'élaboration des produits. Elle permet en effet de protéger ceux-ci, par exemple, des risques de concurrence déloyale ou de contrefaçon. C'est ce contrôle qui donne sa pleine légitimité à l'ensemble de la procédure. Cet amendement tend à intégrer la promotion des produits issus d'exploitations respectueuses de la biodiversité parmi les objectifs de la politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires, et des produits de la mer.

Cet amendement vise à rendre obligatoire, d'ici à cinq ans, l'inscription de critères liés au respect de la biodiversité dans les cahiers des charges des signes de qualité et des mentions valorisantes.

la SNDI, devrait être entérinée au mois de juillet prochain, le concept même de déforestation importée reste à définir. C'est tout l'objet de cet amendement. Nous devons nous emparer pleinement de ce sujet, car ce sont près de 7 millions d'hectares de forêt qui disparaissent chaque année dans les pays tropicaux, et c'est l'agriculture qui reste le principal moteur de la déforestation. Alors que la demande globale pour la production ne cessera d'augmenter, nous sommes persuadés que la sécurité alimentaire pourra être atteinte par d'autres moyens que par l'expansion des zones agricoles au détriment des forêts. Nous devons donc mettre en place un cadre légal et réglementaire efficace pour que nos acteurs prennent leurs responsabilités. En effet, les entreprises françaises figurent parmi les premiers acheteurs de commodités forestières et agricoles ; elles ont par conséquent une responsabilité particulière. Dans le plan Climat publié au mois de juillet 2017, le Gouvernement s'était engagé à « mettre un terme à la déforestation importée ». La France doit être le moteur européen de cette lutte.

le monde sur cette question. Ainsi, la déclaration de New York de 2014 a fixé un objectif de réduction de la moitié du rythme de disparition des forêts d'ici à 2020, mais de fin de leur perte à l'horizon 2030. Hélène Clark, lorsqu'elle a été administratrice du

nous ne souhaitons pas valoriser les produits issus de la déforestation importée. Cela nous ramène au débat que nous avons eu voilà quelques semaines sur la réouverture de l'usine de La Mède et l'importation d'huile de palme.

M. Roland Courteau. Cet amendement vise à poser le principe selon lequel la France devra cesser d'importer des produits contribuant à la déforestation massive dans le monde en 2021. Il s'agit de lutter contre l'abattage des forêts primaires et tropicales qui nuit profondément à l'équilibre de nos écosystèmes. Il convient, d'une part, que la France soit exemplaire dans ce domaine, afin de rendre sa parole audible et crédible à l'étranger, d'autre part, que nous soyons cohérents avec les récentes déclarations du ministre de la transition écologique et solidaire, qui a indiqué vouloir mettre fin à la déforestation importée. Nous avons bien conscience que la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée est en cours d'élaboration et qu'elle sera finalisée à l'été. Toutefois, l'adoption de cet permettrait d'ores et déjà de concrétiser certains engagements forts. À l'instar d'un autre sujet beaucoup plus sensible que nous aborderons tout à l'heure, nous ne comprenons pas pourquoi le Gouvernement refuserait d'inscrire dans son projet de loi

la volonté du Gouvernement. La plupart des entreprises privées visées par la stratégie ont déjà des engagements zéro déforestation pour 2020. Nous proposons par conséquent d'instaurer cet objectif pour le secteur public à puisque la majorité des achats publics sont effectués auprès de ces entreprises. Il existe même déjà des certifications et des démarches certifiées par une tierce partie indépendante permettant de garantir l'absence de déforestation- soja, huile de palme, cacao, noix. L'objectif pour 2025 concerne la conversion d'écosystèmes naturels : conversion de forêts primaires et secondaires, savanes, garrigues et prairies naturelles, tourbières et autres zones humides. Les plantations ne sont pas considérées comme des écosystèmes naturels. Les zones de pâturage destinées au bétail qui sont clôturées ou dominées par une végétation non indigène ne sont pas non plus considérées comme des écosystèmes naturels. Cependant, les systèmes pastoraux ou autres destinés à l'élevage du bétail dans les prairies indigènes sont généralement considérés comme tels. Cet amendement a pour objet de fixer un cap pour 2025 et de laisser suffisamment de temps pour mettre en place les dispositifs permettant d'y parvenir.

de n'acheter que des produits n'ayant pas contribué à la déforestation importée. Cet objectif s'inscrit pleinement dans la lignée du plan Climat, dont l'axe 15 entend interdire l'importation de produits contribuant à la déforestation. Il faut donc que cet objectif s'applique

Il existe des certifications et des démarches certifiées par une tierce partie indépendante permettant de garantir l'absence de déforestation, que ce soit pour le soja, l'huile de palme, le cacao, la noix.

Je rappelle que, en raison de l'adoption de l'article 11 B, nous avons ajouté la promotion des produits n'ayant pas contribué à la déforestation importée à la liste des objectifs de la politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires

? Conformément aux voeux du Président de la République, la France va se doter d'une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Concernant les industries agroalimentaires, il est important de souligner que

Ainsi, en France, une grande entreprise qui produit du pain de mie avec une filière blé 100 % française a supprimé l'huile de palme dans la fabrication de ses produits. Il faut saluer ces gestes environnementaux. Pour autant, aucun instrument européen n'existe aujourd'hui pour certifier que les produits agricoles et alimentaires importés au sein de l'Union européenne sont exempts de déforestation. La France est en train de pousser la Commission européenne pour qu'un plan d'action communautaire soit mis en place. Nous ne pouvons exiger des fournisseurs de l'État français

M. Fabien Gay. Cet amendement vise à inscrire dans le code rural et de la pêche maritime la responsabilité de l'État dans le domaine du respect de la réglementation concernant la chaîne agroalimentaire. En effet, la chaîne agroalimentaire s'est complexifiée et allongée et a une structure hétérogène, puisqu'elle touche à de nombreux métiers. En outre, elle est composée d'acteurs dont la dimension économique et le nombre à chaque échelon sont très disparates. Au sommet se trouvent les consommateurs ; à l'autre extrémité, près de la base, se situent les agriculteurs. Entre ces deux entités, les grandes centrales d'achat des groupes de la distribution ont une taille et un pouvoir économique sans commune mesure du fait de leur concentration.

Cette situation impose donc que l'État puisse jouer un rôle réglementaire pour cette chaîne. C'est le sens de notre amendement. Afin d'aller plus loin, nous proposons d'y associer les laboratoires départementaux d'analyses, ainsi que l'ensemble des acteurs publics et privés contribuant au respect de la législation relative à la chaîne agroalimentaire. Quel

? Cet amendement, mon cher collègue, me semble en partie satisfait puisque l'exploitant doit mettre en oeuvre de suite une procédure de retrait et en informer immédiatement les consommateurs.

n'est pas utile lorsque les produits sont encore sous la responsabilité des opérateurs, ou lorsqu'il s'agit de résultats d'autocontrôle sur l'environnement de production. Une telle information ne manquerait pas de créer un climat anxiogène et d'induire de la confusion chez les consommateurs, alors même que les produits n'ont pas été mis sur le marché.

Cet amendement est important, car il vise à supprimer l'obligation de contre-expertise en cas d'autocontrôle défavorable. Les industriels et les distributeurs ont l'obligation d'informer les services de contrôle dès qu'ils ont connaissance d'un risque pour la santé publique. Les mesures de gestion doivent pouvoir être prises immédiatement après un résultat d'autocontrôle défavorable. La réalisation d'une contre-analyse aurait pour conséquence de retarder la prise de mesures de protection pour la santé publique,

L'amendement n° 188 est de nature à transférer les responsabilités de la sécurité sanitaire de la chaîne alimentaire des exploitants à l'autorité administrative, ce qui contrevient à la réglementation européenne. La commission y est donc défavorable.

Je rappelle qu'un agent pathogène dans l'environnement de production n'induit pas mécaniquement une contamination des produits sortis de l'usine. C'est pourquoi il nous semble nécessaire, monsieur le ministre, de prévoir deux procédures différentes, afin de ne pas déresponsabiliser l'exploitant et de respecter ainsi le droit européen, sans opérer une surtransposition trop forte. Lorsqu'il constate que son environnement de production est potentiellement concerné par la présence d'un agent pathogène, l'exploitant

aura alors l'obligation d'avertir l'autorité administrative d'un risque de contamination de son environnement de production. Revenir sur cette rédaction, c'est imposer une surtransposition forte, en alignant les procédures d'autocontrôle de l'environnement de production sur les procédures d'autocontrôle des produits. Pour toutes ces raisons, la commission émet

Valérie Létard, vise à répondre aux craintes des petits producteurs face à l'afflux des demandes de contrôles et à éviter des traitements différenciés entre les territoires. Il est important de prévoir une demande motivée de la part de l'autorité administrative et surtout de ne pas exclure le producteur du circuit d'information relatif relatif à la communication des résultats des contrôles exercés sur ses propres produits. L'autorité administrative ne peut pas se permettre des contrôles aléatoires et discriminants. En conséquence, l'information qu'elle demande doit être un outil au service d'une gestion de crise avérée, latente ou potentielle.

reviendrait, en n'intégrant pas les producteurs au circuit d'information, à remettre en cause la responsabilité et leur rôle capital de ceux-ci dans la mise en oeuvre de leur maîtrise sanitaire. Un indéniable travail de mise aux normes des ateliers et de formation des producteurs aux questions de sécurité sanitaire est effectué depuis plusieurs années.

le risque n'est pas négligeable, en les déresponsabilisant, de réduire le nombre d'autocontrôles, ce qui serait largement contre-productif et contraire au paquet Hygiène de 2006. Dans l'esprit du paquet Hygiène, l'exploitant est bien responsable de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires qu'il met sur le marché. Dès lors, il paraît normal qu'il soit tenu informé si l'autorité administrative demande, dans le cadre d'un contrôle officiel, un résultat d'analyse. La commission est donc favorable à

Cet amendement tend donc à mettre l'accent sur les audits en matière de bonnes pratiques de fabrication, d'hygiène et de respect des principes HACCP mis en place par le fabricant sur ses chaînes de production, ses locaux, son environnement immédiat, ses matières premières et son personnel. Le ministre de l'économie et des finances ayant affirmé qu'il n'y aurait pas d'augmentation du nombre de personnels qualifiés dans les services de contrôle, en particulier dans les directions départementales de la protection des populations, cet amendement tend à modifier les modes de contrôle de ces services.

Cet amendement vise à renforcer l'information du consommateur en cas de crise sanitaire liée à des denrées alimentaires. Il s'agit de permettre à chaque citoyen, de façon rapide et claire, d'avoir accès à l'ensemble des informations.

? Cet amendement ne vise que les décisions de retrait prononcées par l'autorité administrative, alors que ces décisions peuvent, nous le savons, être aussi prises par les fabricants de produits

est vrai que nous devons tirer les leçons de la récente crise chez Lactalis. Le ministère de l'économie et des finances, dans le cadre du Conseil national de la consommation, a engagé des réflexions sur les procédures de retrait et

à l'industriel d'apporter la preuve que le produit qu'il met sur le marché ne présente aucun danger particulier pour les consommateurs.

Cet amendement tend ainsi à imposer aux professionnels la réalisation d'un état chiffré des produits retirés ou rappelés. Cette traçabilité permettra de renforcer la gestion des opérations par les professionnels et leur contrôle par les services de l'État. Le non-respect sera pénalement sanctionné, dans le code de la consommation pour les denrées végétales et dans le code rural et de la pêche maritime pour les denrées animales. Nous proposons, par ailleurs, de maintenir l'actuel régime de sanction délictuelle pour les producteurs et importateurs,

que ce soit les producteurs, les transformateurs ou les distributeurs, assurent des procédures de retrait et de rappel publiques immédiatement, dès que la sécurité des produits est mise en doute. Si, comme

lait avaient été produits en octobre 2017, il a fallu attendre cinq mois et un contrôle de la direction départementale de la protection des populations de Vendée avant qu'ils soient rappelés.

un avis favorable sur l'amendement du Gouvernement qui reprend les éléments issus du travail de nos commissions. Nous serons particulièrement attentifs, monsieur le ministre, à la mise en place du régime contraventionnel

L'article L. 411-1 du code de la consommation prévoit en effet une obligation d'autocontrôle lors de la première mise sur le marché d'un produit ou d'un service. Cependant, aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect de cette obligation. Le présent amendement tend donc à modifier l'article L. 451-1 du code précité relatif aux sanctions en cas de manquement à l'information du consommateur pour remédier à ce vide juridique. ? Il existe déjà un certain nombre de sanctions. En particulier, si les autocontrôles ne sont pas effectués conformément à ce qui est prévu dans le plan de maîtrise sanitaire de l'établissement,

La publication des résultats des opérations de contrôle sanitaire est une démarche d'ores et déjà inscrite dans le droit français. Le décret du 15 décembre 2016 a ainsi créé les articles D. 231-3-8 et D. 231-3-9 du code rural et de la pêche maritime qui précisent les modalités de publication des résultats des contrôles. En outre, l'arrêté du 28 février 2017, relatif aux modalités d'application du décret susmentionné, a renforcé ces prérogatives de publication des résultats de contrôle. Si l'application de la loi d'avenir pour l'agriculture, a permis la mise en place du dispositif Alim'confiance, site permettant d'accéder aux informations relatives aux contrôles officiels en matière de sécurité sanitaire des aliments, ce dispositif n'est pas exempt de critiques informations cantonnées aux questions d'hygiène des aliments, sans mention de la qualité, de la sécurité ou des règles d'information, suppression des informations postées après un an sur le site, etc.

publiés sur le site internet Alim'confiance, que je vous invite une nouvelle fois à télécharger. Le dispositif étant récent, il peut effectivement être amélioré. Les services y travaillent, à ma demande. Par conséquent, il est prématuré aujourd'hui d'étendre le dispositif à d'autres critères d'appréciation, voire à d'autres produits, avant

Les crises sanitaires et médiatiques, notamment celle de Lactalis, ont révélé un besoin de laboratoires accrédités et indépendants sur l'ensemble du territoire. Il est préférable de confier les autocontrôles à des laboratoires accrédités, afin de viser un haut niveau d'exigence technique et une homogénéité des prestations entre laboratoires. La même exigence devra être imposée aux laboratoires chargés par les autorités sanitaires de vérifier et de contrôler les autocontrôles. À cet égard, monsieur le ministre, les laboratoires départementaux d'analyses rappellent qu'ils assument aujourd'hui une large mission d'épidémiosurveillance sur le territoire national dans les domaines de la santé animale, de l'hygiène alimentaire, de la santé des végétaux et de la surveillance sanitaire des produits de la mer. Leur indépendance, leur répartition sur l'ensemble du territoire et leur haut niveau d'expertise analytique sont des garanties de réactivité et d'expertise en matière de sécurité sanitaire. À ce titre, ils contribuent largement au maillage sanitaire français dont bénéficient les acteurs des filières de production, grâce au soutien financier des collectivités locales, qui assurent ainsi leurs missions d'épidémiosurveillance. C'est la raison pour laquelle les élus départementaux souhaitent que ces laboratoires soient préservés sur l'ensemble du territoire. Quel est l'avis de la commission

bien évidemment le cas des laboratoires d'analyses départementaux, qui ne sont pas concernés par cet article. L'autre niveau, qui, lui, est visé par cet article, regroupe les laboratoires réalisant des autocontrôles qui ne sont généralement pas des laboratoires effectuant des contrôles officiels et qui ne suivent aujourd'hui aucune procédure d'accréditation ou de comparaison interlaboratoires. L'article 11 A renforce la réglementation pour ces laboratoires, en prévoyant qu'ils réalisent des autocontrôles. Il ne supprime donc pas l'accréditation officielle, mais en ajoute une, au bénéfice de la sécurité des consommateurs. L'amendement qui nous est proposé tend à accréditer tous les laboratoires accomplissant des autocontrôles. Son adoption poserait deux difficultés part, cette transposition structurelle de la réglementation européenne aura des surcoûts importants pour l'ensemble des entreprises agroalimentaires ; d'autre part, compte tenu de la situation financière de nombreux laboratoires,

Les restrictions prises sur le dioxyde de titane sont une avancée, que nous saluons et qui ne doit pas s'arrêter à la seule question de l'agroalimentaire. L'additif E171 est pointé du doigt depuis de nombreuses années, et les études menées ne manqueront sans doute pas d'attester son potentiel toxique pour l'organisme et son franchissement des barrières biologiques chez l'homme. Le dioxyde de titane ne sert à rien d'autre qu'à blanchir. Il n'apporte rien de plus. L'enjeu sanitaire concerne en premier lieu les enfants, amateurs de confiseries. Au-delà de l'exemple du dioxyde de titane, qui est emblématique, nous devrions dès à présent nous interroger sur l'ensemble des additifs alimentaires, notamment quand ces substances ont pour seule fonction de colorer, blanchir ou modifier le goût des aliments. Un projet ambitieux pour une loi sur l'alimentation saine et durable aurait été de lancer une véritable réflexion dépassant le seul cadre du dioxyde de titane je pense bien évidemment, tout comme Angèle Préville, à l'ensemble des substances chimiques nocives ajoutées aux denrées alimentaires et aux produits transformés dont les risques pour la santé sont avérés. Je conclus ce propos

milliers de médicaments vendus aujourd'hui en France contiennent du E171. Le retrait du dioxyde de titane sera-t-il également imposé à

qu'il ne puisse être lu comme une injonction du Parlement au Gouvernement. Nous ne sommes qu'au début du travail, mais nous avons fait une belle avancée avec la suppression du dioxyde de titane dans un certain nombre

Cette proposition ne modifie pas le fond de l'article, qui prévoit une suspension de la mise sur le marché du dioxyde de titane comme additif alimentaire et des denrées alimentaires en contenant. En commission, nous avons bien évidemment pleinement soutenu cette mesure, compte tenu des risques associés à cette substance, qui est d'ailleurs utilisée à des fins purement esthétiques dans l'alimentation. Un avis rendu par le Haut Conseil de la santé publique ce lundi 25 juin nous conforte dans cette décision, en mettant en évidence les risques du dioxyde de titane lorsqu'il est utilisé sous forme nanoparticulaire, ce qui est le cas.

Je profite de l'occasion pour souligner qu'un usage approprié du principe de précaution, lequel justifie cette suspension, implique une concertation avec les parties prenantes, en l'occurrence les producteurs, distributeurs et utilisateurs du dioxyde de titane, pour leur donner de la visibilité, afin de leur permettre de réorganiser leurs activités À ce titre, monsieur le ministre, pouvez-vous nous apporter des éléments sur le calendrier de cette procédure de suspension ? Par ailleurs, le Gouvernement a-t-il déjà eu des échanges avec les acteurs du secteur ou des rencontres sont-elles prévues prochainement à ce sujet ? La parole

ministre. Monsieur le rapporteur pour avis, vous m'avez interrogé sur les prochaines étapes de la procédure de suspension du dioxyde de titane et sur les conditions dans lesquelles les acteurs du secteur, les producteurs, les distributeurs et les utilisateurs, ont été ou seront consultés ou associés à cette

monsieur le ministre, mes chers collègues, lors de la discussion du projet de loi de modernisation de notre système de santé, en 2016, j'avais tenté d'imposer aux industriels de l'alimentation des objectifs clairement établis concernant la qualité nutritionnelle de leurs recettes manufacturées.

de matières grasses totales, d'acides gras saturés, de sucre ou de sel. Pis, les aliments ultratransformés se retrouvent partout dans les rayons, avec des taux en sucre ajouté et en sel très importants.

pour laquelle ont été décryptés les ingrédients de cent denrées alimentaires. Croisée à une série d'études internationales, notamment celle de la revue qui a été publiée de l'année, elle semble établir un lien sérieux entre nourriture ultratransformée et risque de cancer. Un autre problème de santé majeur en découle, considéré comme un véritable fléau par l'Organisation mondiale Un Français sur deux est en surpoids, quand 15,8 % des hommes et 15,6 % des femmes sont atteints d'obésité. Fait plus grave, le taux de personnes en surcharge pondérale- surpoids plus obésité -s'élève, au total, à 56,8 % pour les hommes et à 40 % pour les femmes. Malgré les efforts consentis depuis plusieurs années et les différentes campagnes de sensibilisation, cette pathologie est très prégnante aux Antilles, où elle touche toutes les générations. En 2014, 4,8 % des enfants des classes maternelles et 5,5 % des enfants des classes de CM2 les départements d'outre-mer souffraient d'obésité. N'oublions pas également que l'une des conséquences de ce fort taux d'obésité est l'augmentation des cas d'AVC et des maladies cardiovasculaires sur notre île. C'est pourquoi

produite localement, notamment en direction de notre jeunesse, pour tout ce qui concerne la restauration scolaire. Cependant, il est évidemment nécessaire de prévoir un dispositif de suivi pour pouvoir suivre l'avancée de cette mesure et voir si l'on atteint nos objectifs, pour que l'orientation que nous avons inscrite dans ce texte ne reste pas sans concrétisation sur le terrain. L'amendement du rapporteur qui a été adopté hier répond partiellement à cet objectif, en créant, à l'échelon régional, une instance de concertation sur l'approvisionnement de la restauration collective.

qui vise à étendre les missions de l'Observatoire de l'alimentation au suivi des données qualitatives et quantitatives relatives à la restauration collective responsable. Ainsi,

L'Observatoire pourrait éventuellement prendre le nom d'« observatoire de l'alimentation et de la restauration collective responsable ». Il nous permettrait de rendre opérationnels les objectifs que nous inscrivons dans la loi et qui doivent être une priorité, mais aussi de valoriser les expériences réussies, notamment les modèles économiques performants pour accompagner les gestionnaires de la restauration collective, particulièrement les petites collectivités locales. Quel est l'avis de la commission

du Gouvernement ? Monsieur le sénateur, il n'est pas souhaitable de confier à l'Observatoire de l'alimentation la mission de veiller au respect de l'obligation prévue à l'article 11 du projet de loi, parce qu'il n'en a pas les moyens. De manière générale, il faudra prévoir les

les travaux conjoints de l'INRA et de l'ANSES, au sein de l'Observatoire de la qualité de l'alimentation, montrent qu'il n'y a pas eu de diminution significative de la consommation de matières grasses totales, d'acides gras saturés, de sucre ou de sel. à ces chiffres, vise à ce que soient mis en place des objectifs ambitieux, portant sur l'ensemble des produits des filières directement responsables de ces déséquilibres alimentaires. En outre, son adoption constituerait un levier important pour incorporer une part accrue de matières premières agricoles à valeur nutritionnelle significative dans la fabrication des produits alimentaires. D'ailleurs, dans son avis sur l'actualisation des repères du programme national nutrition santé, l'ANSES défendait une position proche de cette demande, en proposant que les pouvoirs publics soient chargés de déterminer un objectif chiffré de diminution des taux de sucre par famille d'aliments. Cette mesure serait assortie d'un calendrier permettant de fixer des délais à respecter pour chaque objectif.

fixe des objectifs clairs en matière de réduction des taux de matières grasses, de sucre et de sel par famille de produits alimentaires. Il s'agit bien entendu de répondre à l'explosion du phénomène d'obésité en France, particulièrement chez les jeunes, en renforçant le rôle stratégique de l'État dans ce domaine.

l'article L. 230-4 du code rural et de la pêche maritime prévoit que l'État incite les opérateurs du secteur agroalimentaire à mettre en oeuvre des accords collectifs ayant pour but d'améliorer la qualité nutritionnelle des denrées alimentaires. Pour ce faire, ces opérateurs fixent eux-mêmes, à ce jour, des objectifs à atteindre, conformément aux orientations définies dans le PNNS. L'amendement que nous vous proposons vise à renforcer ce afin que les acteurs de la chaîne alimentaire soient contraints d'y intégrer des objectifs clairs, permettant de procéder à des évaluations avec les partenaires.

De nombreux rapports d'observations de l'Observatoire de la qualité de l'alimentation, de l'ANSES et de l'INRA pointent du doigt le manque de baisse significative des consommations de matières grasses totales, d'acides gras saturés, de sucre ou de sel. Dans son avis de décembre 2016, l'ANSES proposait déjà de réactualiser les repères du programme national nutrition santé et demandait que les pouvoirs publics soient chargés de déterminer un objectif de

des États généraux de l'alimentation et du plan national de santé publique diffèrent de celles qui sont ici proposées. Nous souhaitons donner un nouvel élan aux engagements des professionnels en privilégiant des approches ambitieuses mesurables et vérifiables. La fixation de seuils réglementaires interviendra

Disons plutôt qu'on a manifesté une nouvelle espérance vis-à-vis de l'industrie agroalimentaire. Malheureusement, neuf mois après

Des recherches récentes montrent que la consommation régulière de ces aliments recomposés, souvent riches en sucres et en graisses, favorise l'apparition de maladies métaboliques chroniques, comme le diabète, l'hypertension ou l'obésité.

l'alimentation. Avec le manque d'activité physique, l'alimentation est un élément déterminant de l'émergence des principales pathologies chroniques- cancer, diabète ou maladies cardiovasculaires le schéma régional de santé comporte des volets consacrés à l'offre de soins, à l'accès aux soins, à la sensibilisation de la population et des professionnels aux maladies vectorielles, ou encore à des besoins spécifiques liés à la situation géographique. Le lien entre santé et alimentation étant extrêmement fort, nous proposons que chaque schéma régional de santé intègre demain un volet consacré à l'alimentation, notamment en termes de sensibilisation de la population et d'éducation aux bonnes conduites alimentaires auprès des plus jeunes.

Il classe en cinq catégories, allant de A au E et du vert au rouge, les produits alimentaires en fonction de leurs qualités nutritionnelles. Ainsi, les produits riches en nutriments à favoriser, comme les fibres, les protéines, les fruits et les légumes, obtiendront un score plus proche du vert et du A, et ceux qui sont riches en nutriments à limiter- sel, sucres et gras -un score plus proche du rouge et du E. Cette information transparente et directe vise, d'une part, à mieux informer le consommateur dans ses choix et, d'autre part, à terme, à inciter les industriels à améliorer la composition et la qualité nutritionnelle de leurs produits. Des études menées par les autorités sanitaires ont démontré que le logo Nutri-score orientait le choix des consommateurs, en particulier les plus jeunes, Si la mention du Nutri-score sur les emballages n'a pas de caractère obligatoire pour des raisons de conformité au droit européen, la présence de ce logo est néanmoins recommandée par les autorités. Un certain nombre d'entreprises s'est engagé à le faire figurer sur une partie de ses produits. Les avancées dans ce sens s'avérant encore insuffisantes, le présent amendement vise à rendre obligatoire la mention du Nutri-score sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires.

et activités promotionnelles, directes ou indirectes, portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés destinés aux mineurs sont interdits, sur tous supports audiovisuels, radiophoniques, ou électroniques. Dans un rapport de 2016, l'Organisation mondiale de la santé soulignait les effets néfastes du marketing d'aliments hautement énergétiques, riches en matières grasses, en sucre ou en sel sur les enfants, lequel entraîne une propension à préférer les aliments et modes d'alimentation peu sains et favorisant l'obésité. J'ai déjà souligné qu'il

à renforcer la protection des enfants et des adolescents par l'encadrement très strict de la publicité en faveur des produits à forte teneur en sucres ou en matières grasses. On se doit de favoriser la qualité de l'alimentation de nos enfants

Nous savons que cette proposition a déjà été rejetée à plusieurs reprises, mais nous la maintenons, car nous la jugeons opportune. Il est inutile de rappeler l'influence de la télévision, de la radio, des médias, surtout chez les plus jeunes enfants. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons réellement agir sur les conduites alimentaires. mettre de côté la problématique de la publicité. En outre, l'interdiction que nous proposons complétera utilement les dispositions de la loi du 20 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique. Je précise que le II de notre amendement permettra,

Des données incontestables montrent que la commercialisation d'aliments nocifs pour la santé et de boissons sucrées a un lien avec l'obésité de l'enfant ». Elle ajoute : : « Même si l'industrie déploie un nombre croissant d'initiatives volontaires, l'exposition à la commercialisation des aliments nocifs pour la santé reste un problème majeur appelant un changement pour protéger tous les enfants de façon égale. La volonté de corriger l'augmentation continue des cas d'obésité de l'enfant devrait donc tendre à réduire l'exposition des enfants à la commercialisation des aliments nocifs pour la santé. Actuellement, la France la France se contente des engagements volontaires de l'industrie agroalimentaire sur le marketing ciblant les enfants, comme le. De nombreuses études ont montré que ces engagements volontaires étaient très insuffisants, voire inopérants, pour assurer une prévention efficace de marketing ciblant les enfants pour des aliments déséquilibrés. La nécessité de « limiter l'influence de la publicité et du marketing alimentaire sur les enfants en les réglementant et [d']encadrer la promotion des marques associées à des aliments peu favorables au plan nutritionnel » est aujourd'hui inscrite

n° 326 rectifié. Cet amendement vise à encadrer le marketing alimentaire à destination des mineurs sur internet. Les effets néfastes des publicités pour des aliments peu sains sont rappelés par l'OMS depuis plusieurs années. Il est aujourd'hui indispensable de dupliquer l'encadrement existant et les médias délinéarisés, par lesquels les jeunes publics sont de plus en plus attirés. Ainsi, il est proposé que les jeux, applications et sites internet portant sur ce type de produits ou utilisant leur logo ou mascotte ne puissent être accessibles aux mineurs.

-ou des logos évoquant clairement le type de produits en question, tel l'animal d'une marque de céréales. Ainsi, si l'aliment n'est pas le sujet principal du jeu, la mascotte relève clairement de la publicité et aura forcément tendance à attirer l'enfant vers le produit qu'elle représente.

Depuis plusieurs années, l'OMS tire la sonnette d'alarme et appelle à limiter les effets néfastes, auprès du grand public, des publicités pour des aliments peu sains. Il paraît aujourd'hui indispensable de mettre en place un encadrement sur internet et les médias délinéarisés, dont les jeunes publics sont de plus en plus friands. Ainsi, nous proposons que les jeux, applications et sites internet portant sur ce type de produits ou utilisant leur logo ou mascotte ne puissent être accessibles aux mineurs. En plus d'éviter que ce jeune public ne soit attiré sur des sites vantant les mérites d'une alimentation déséquilibrée, l'adoption de cet amendement permettra d'empêcher tout contournement, à créer des divertissements reprenant des mascottes et/ou des logos qui évoquent clairement ce type de produits, tel l'animal d'une marque de céréales. Ainsi, si l'aliment n'est pas le sujet principal du jeu, la mascotte relève clairement de la publicité et aura tendance à attirer l'enfant vers le produit qu'elle représente.

serait rejeté. Nous connaissons l'argument du Gouvernement, qui revient à considérer qu'il appartient à la charte alimentaire du CSA d'aborder la question de la limitation ou de l'encadrement de la publicité en faveur de certains produits manufacturés. Par ailleurs, nous avons bien pris connaissance de la deuxième charte alimentaire du CSA, signée en 2013, qui comporte un volet visant à promouvoir une alimentation saine et une activité physique. Cependant, outre le fait que cette charte, selon nous, ne va pas suffisamment loin, nous considérons que, sur des questions de cette importance, il est fort regrettable que les législateurs que nous sommes soient ainsi exclus du processus décisionnel. De plus, il s'agit ici d'une question de santé publique. Je ne vois pas en quoi le CSA serait plus compétent que le Parlement pour l'aborder. En tout état de cause, par cet amendement, nous demandons que le Gouvernement remette un rapport au Parlement, afin de préciser concrètement les engagements qu'il compte prendre dans la future charte alimentaire pour encadrer et limiter la publicité de certains produits alimentaires à destination des plus jeunes.

, 606 rectifié et 679 rectifié ils concernent uniquement les jeux, applications et sites internet, qui ne pourraient faire référence à des produits alimentaires qu'auprès des majeurs.

Je veux également insister sur l'ensemble des instruments existants pour réguler aujourd'hui la communication alimentaire auprès des jeunes. Ainsi, la loi de décembre 2016 a supprimé, le 1 janvier de cette année, la publicité commerciale à destination des enfants de moins de douze ans dans les émissions destinées à la jeunesse. Par ailleurs, la charte du Conseil supérieur de l'audiovisuel comporte des dispositions en la matière. Il est prévu, monsieur le ministre, de la renforcer dans les prochains mois,

nous considérons que les pouvoirs publics et le CSA, l'organe régulateur, sont suffisamment mobilisés sur ce sujet qui ne justifie pas un nouveau rapport. La commission y est donc défavorable. ? Sur ces sujets, nous l'avons toujours dit, nous privilégions le travail avec le CSA sur la charte de régulation. Le CSA est

Ces aliments présentent des risques de carence et de déséquilibres pondéraux pour la santé lorsqu'ils sont consommés avec excès. Ils entraîneraient diabète, surpoids ou obésité, maladies cardiovasculaires et AVC précoces, ou encore hypertension artérielle. Les experts prévoient même que les enfants d'aujourd'hui pourraient être la première génération à avoir une moins bonne santé et une durée de vie plus courte que leurs parents. Selon l'OMS et l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, les publicités télévisées influenceraient les demandes d'achats alimentaires et les habitudes de consommation des enfants, cibles privilégiées des publicitaires puisqu'ils sont à la recherche constante de modèles auxquels s'identifier. Selon l'UFC-Que Choisir, les enfants les plus exposés aux publicités sont aussi ceux qui consomment le plus de produits gras et sucrés. Un enfant qui regarde les publicités lui étant destinées ingère 300 calories de plus par jour. De la même manière, 76 % des demandes d'achats des enfants de quatre à dix ans sont en lien avec une publicité, et 82 % des enfants demandent à leurs parents des produits qu'ils ont vus à la Cet amendement vise ainsi, selon les recommandations de l'OMS de 2010, à réduire l'exposition des enfants à la promotion d'aliments manufacturés nocifs, afin d'encourager une alimentation saine, ce qui est d'ailleurs l'un des objectifs de la stratégie nationale de santé pour Face à ce problème sociétal, nous nous devons d'être ambitieux. Se reposer sur les engagements volontaires des industriels ou sur les responsabilités des parents face à l'éducation alimentaire de leurs enfants ne suffira pas. Ce qu'il faut, c'est réguler l'environnement des enfants. Même si le rôle de l'éducation parentale reste important, ce sont généralement les enfants qui sont prescripteurs d'achats, puisque 87 % d'entre eux disent obtenir ce qu'ils demandent. Ce phénomène de socialisation inversée, dans lequel les décisions économiques de la famille sont dévolues aux enfants, suggère qu'il sera inévitable de mettre des limites à la publicité pour protéger la santé de nos enfants.

Il prévoyait notamment que les actions en matière de lutte contre la précarité alimentaire et en faveur du respect du bien-être animal et d'une alimentation responsable, équitable et durable soient intégrées dans le extrafinancier. Le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, dit

Elle ne peut se résumer à son objectif de maximisation de profits, mais doit intégrer les dimensions environnementales, sociétales et sociales. La responsabilité sociale des entreprises permet d'intégrer les préoccupations sociétales dans les activités économiques de nos sociétés et dans leurs interactions avec l'ensemble des parties prenantes. Par cet amendement, nous souhaitons souligner, à l'intérieur même du dispositif de RSE, les engagements sociétaux de nos entreprises en faveur du don alimentaire, du respect du bien-être animal et d'une alimentation durable. Ce dispositif permet donc de mettre en place un levier d'action pour améliorer concrètement les conditions de vie des animaux, lutter contre la précarité alimentaire ou encore défendre une alimentation durable. Il permettra à tout citoyen, dans ses statuts de collaborateur, de consommateur ou d'épargnant, de procéder à une comparaison des performances des entreprises en la matière.

doit être clairement encadrée. Dans ce cadre, il est important de protéger efficacement les données personnelles de nos concitoyens, y compris de nos agriculteurs. Ainsi, il n'est pas concevable que les bases de données de l'État, qui rassemblent des données personnelles des agriculteurs, puissent être transmises à des organismes privés, y compris interprofessionnels : à l'heure actuelle, la gouvernance, la représentativité et les pratiques de ces organismes ne permettent pas de donner les garanties suffisantes pour une utilisation respectueuse des principes les plus fondamentaux de la protection des données individuelles. C'est dans cette logique que nous vous proposons, par cet amendement, de supprimer cet article. La parole En effet, cet article permet à l'État de recourir à des opérateurs privés pour la collecte et le traitement des données, ainsi que pour des informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers sanitaires. Cette possibilité, qui est d'ailleurs déjà utilisée en matière d'identification des animaux, devrait permettre,

mais à agréer un dispositif de collecte et de traitement de l'information à caractère réglementaire. Une telle disposition, qui existe en matière d'identification des animaux, a montré toute sa pertinence. Il s'agit de dupliquer, pour ce qui nous concerne, certaines données réglementaires à caractère sanitaire, liées notamment à l'influenza aviaire. Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces amendements

est actuellement engagée entre les États membres et la Commission européenne. Il s'agit bien entendu d'une compétence européenne, mais qui a des impacts extrêmement importants pour l'agriculture française. Aussi, il paraît indispensable que le Gouvernement puisse présenter sa stratégie en la matière devant la représentation nationale. Pour l'heure, les communications émanant du ministère de l'agriculture ne présentent pas une vision claire et lisible des arbitrages déjà rendus ou des perspectives visées pour la période 2021-2027. Par cet amendement, il s'agit d'obtenir une présentation axée autour de trois objectifs essentiels pour le développement et l'avenir de l'agriculture française : un renforcement du couplage des aides ; l'introduction de mécanismes « contracycliques » destinés à amortir les chocs liés à l'évolution des cours mondiaux des denrées agricoles et la mise en place d'un plafonnement, de manière à éviter la captation des aides agricoles par les structures les plus importantes, qui bénéficient de gains de productivité liés à leur taille et à leur éventuelle emprise sur le marché. Quel est l'avis de la commission

Les débats ont d'ailleurs permis au Gouvernement de préciser ses orientations. Le Sénat poursuivra ses travaux. Aux termes de l'article 88-4 de la Constitution, le Gouvernement doit soumettre au Parlement tous les projets d'actes législatifs européens. Le Parlement sera donc associé au déploiement du nouveau cadre de la PAC. Il y sera-

les différents acteurs d'un territoire autour de la question de l'alimentation. Les PAT visent à construire des circuits alimentaires de proximité prenant en compte les dimensions sociales, environnementales, économiques et de santé de ce territoire.

On a beaucoup parlé de répartir la valeur entre les acteurs de la chaîne alimentaire et des difficultés pour y parvenir et garantir un revenu à nos producteurs. Il existe une solution à exploiter : court-circuiter les gros acteurs de l'aval, en relocalisant l'alimentation et en limitant le nombre d'intermédiaires.

avec des déclinaisons dans les EPCI ou les départements de la région. Il y a un certain nombre de formules de périmètres sur lesquelles vous pouvez travailler. En rendant obligatoire la signature de PAT, nous

Cet amendement vise à garantir la qualité des produits vendus aux consommateurs. Face à la multiplication des ventes au déballage sur une partie du territoire national, il est devenu urgent de renforcer la législation actuelle pour garantir la sécurité sanitaire des consommateurs et lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Nombre de ventes au déballage de produits alimentaires frais ou non transformés, essentiellement des fruits et légumes, sont effectuées dans des conditions ne respectant nullement les règles les plus élémentaires d'hygiène et de traçabilité. Régies sous l'empire du régime déclaratif, les ventes au déballage prolifèrent.

un avis défavorable sur cet amendement. Le code de commerce restreint déjà les conditions de vente au déballage, y compris pour les fruits et les légumes frais. Cette vente ne peut pas excéder deux mois, que ce soit dans un même local, sur un même emplacement où dans un même arrondissement départemental. L'adoption de cet amendement conduirait à pénaliser l'ensemble des vendeurs, même ceux qui commercialisent en toute bonne foi, ce qui serait contraire au principe de proportionnalité, sans pour autant pénaliser ceux qui voudraient contourner le code de commerce. Nous devons évidemment

Il s'agit, avec les moyens de contrôle de la DGCCRF, d'essayer de circonscrire au maximum de telles pratiques et d'encourager les pratiques vertueuses ; je pense à ceux qui « payent patente » et à ceux qui sont dûment inscrits au registre du commerce et qui ont la capacité de vendre les produits.

est ainsi libellé : La parole est à M. Jean-Claude Tissot. La demande sociétale pour une alimentation de qualité relocalisée, source de lien social entre producteurs et consommateurs, et produite par des paysans correctement rémunérés et ancrés dans leurs territoires n'a jamais été aussi forte. Les marchés communaux pourraient constituer un puissant levier pour encourager cette dynamique, en incluant, dans les règlements de marché, des moyens de valoriser les étals des producteurs locaux de denrées alimentaires : label, affichage, emplacements réservés, De la même manière que l'article L. 611-8 du code rural et de la pêche prévoit la création de magasins de producteurs dans « une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir », les marchés communaux pourraient distinguer les producteurs agricoles locaux. Certaines communes affichent déjà des politiques très volontaristes pour favoriser l'accès des producteurs aux marchés de plein vent. Cette démarche pourrait être soutenue et encouragée en vue d'une généralisation si les consommateurs pouvaient être avisés de la composition des marchés qu'ils fréquentent. Les amendements

relocalisée, source de lien social entre producteurs et consommateurs et produite par des paysans correctement rémunérés et ancrés dans leur territoire. Les marchés communaux peuvent constituer un puissant levier pour encourager cette dynamique. Nous voulons inclure dans les règlements de marché des critères de priorité pour les producteurs locaux dans l'attribution des emplacements vacants des marchés. Certaines communes affichent déjà des politiques très volontaristes

Cet amendement vise donc à demander au Gouvernement d'apporter une information précise au Parlement sur l'évolution des aides en faveur de l'agriculture biologique, notamment à la lumière du désengagement de l'État concernant les aides au maintien. Quel est l'avis de la commission

des réponses structurelles pérennes à des problèmes profonds qui touchent notre agriculture, il va falloir procéder et raisonner autrement